d’observation ?… Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage. J’informe le Sénat qu’ont été publiées des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, du projet de loi organique relatif à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et du projet de loi relatif à l’industrie verte.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 L’ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission des affaires européennes et de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et Conformément aux articles 8, 8 et 73 du règlement, les listes des candidats remises par les présidents des groupes ont été publiées. Ces listes seront ratifiées s’il n’y a pas d’opposition dans le délai d’une heure.

La séance est levée.